Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je suis très heureuse que nous ayons ce débat aujourd'hui. Il nous offre l'occasion de revenir sur les nombreux textes adoptés en matière de justice et de sécurité durant cette législature. Pêle-mêle, je citerai la loi Asile et immigration, la loi Sécurité globale ou encore les lois sur les violences sexuelles et sexistes et sur les violences sexuelles sur mineurs, toutes accueillies plus ou moins chaleureusement, mais qui prouvent une volonté de réforme, appuyée par une hausse des crédits, qu'il convient de saluer.

des mineurs. Ces mesures, qui permettent notamment une évaluation de la personnalité d'un mineur en difficulté, de sa situation familiale et sociale, de ses conditions de vie et celles de ses parents, sont actuellement réalisées en seize jours en moyenne.

elle permet le jugement rapide des mineurs ayant des antécédents judiciaires. Cette mesure entraîne une augmentation du nombre de condamnations à des peines d'incarcération, ce qui vient conforter le taux particulièrement élevé d'incarcération des mineurs dans notre pays.

la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature, Chantal Arens -en recrutant des magistrats et des greffiers, si possible titulaires. Dépenser mieux enfin pour rendre notre justice plus rapide et plus efficace, pour rétablir la confiance de nos concitoyens et alléger le travail des services de police et de gendarmerie, car l'une ne va pas sans l'autre. Il nous faudrait d'ailleurs réfléchir à la réponse pénale que nous souhaitons apporter,

nombre d'entre nous ont été confrontés à des maires qui, faute d'effectifs de police nationale suffisants, ont créé ou renforcé les effectifs de police municipale, quand bien même cette dernière ne répond pas aux mêmes besoins, ne remplit pas les mêmes missions et ne dispense pas la même formation.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cinq minutes ne suffiront pas à dresser un bilan exhaustif de l'action du Gouvernement en matière de justice et de sécurité, mais je reviendrai sur les principaux textes qui ont marqué ce quinquennat.

(SILT) en 2017, puis la loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, dite SILT 2, de juillet dernier, nous ont démontré le contraire : non seulement toutes les mesures ont été prorogées, mais elles ont également été durcies avec, par exemple, la généralisation des assignations à résidence « déguisées » et celle des perquisitions contrôlées par l'administration, tout en contournant la procédure judiciaire et les droits de la défense. Ce gouvernement a fait le choix d'opérer un tournant radical en matière de police administrative, inspiré par un principe de précaution incompatible avec nos principes démocratiques fondés sur un droit pénal d'interprétation stricte. En matière de renseignement, ce gouvernement a légalisé et étendu des techniques de surveillance intrusives, là encore en maintenant à distance l'autorité judiciaire. Notre pays s'est doté d'un arsenal de surveillance de masse, alors même qu'il disposait déjà d'une législation répressive substantielle. Un virage assez spectaculaire a également été pris avec la loi Sécurité globale, heureusement retoquée pour l'essentiel par le Conseil constitutionnel, mais dont des mesures

et de contrôle des populations. En outre, la loi Sécurité globale est venue renforcer la confusion des genres entre la police nationale, la police municipale, dont les agents reçoivent des prérogatives judiciaires sans la formation nécessaire, et les sociétés de sécurité privée, auxquelles sont délégués des pouvoirs de plus en plus étendus, notamment en matière de terrorisme- elles sont autorisées, par exemple à effectuer des fouilles. J'en viens maintenant au second thème de ce débat : la justice.

alors que des milliers de policiers, massés devant le Palais-Bourbon, réclamaient une réponse pénale plus ferme, le secrétaire général du syndicat Alliance scandait : « Le problème de la police, c'est la justice ! L'indignation parmi les magistrats et le malaise dans la classe politique n'auront pas eu raison du Gouvernement, puisque le garde des sceaux a décidé de répondre à ces pressions en intégrant dans l'urgence,

la limitation des réductions de peine pour les agresseurs de forces de l'ordre. Des mesures purement démagogiques, en parallèle à d'autres prises antérieurement, et pour l'essentiel dans la droite ligne de la réforme de Mme Belloubet, l'ancienne garde des sceaux. La myriade d'articles protéiformes de ces deux lois structurantes de ce quinquennat répond à un objectif dangereux, qui consiste à redresser la justice comme s'il s'agissait de n'importe quel autre service public, en traitant l'embolie diagnostiquée de nos juridictions à coups de mesures gestionnaires et comptables. C'est de l'apogée de cette gestion dont il est question dans la tribune historique des 3 000 magistrats, qui dénoncent « une logique de rationalisation qui déshumanise et tend à faire des magistrats des exécutants statistiques ». Car aussi régalien soit-il, le ministère de la justice n'est pas épargné par la main invisible de Bercy, téléguidée depuis l'Élysée, voire depuis Beauvau. Pour en revenir au présent débat, le Beauvau de la sécurité est assez révélateur de la vision du Gouvernement en matière de sécurité et de justice : « Intérieur et justice unis contre l'insécurité et l'impunité », titre le site du Gouvernement sur le sujet Le débat théorique autour de l'opposition entre efficacité sécuritaire et garantie des libertés individuelles semble désormais dépassé. Les plateaux de la balance ont basculé et les dommages pour notre État de droit sont importants. Voilà pour nous le triste bilan du Gouvernement en la matière.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette fin d'année 2021 coïncidant avec la fin du quinquennat, la période est particulièrement propice aux bilans. aux bilans. Nous parlons ce soir de justice et de sécurité, deux thèmes que les commentateurs de tous bords ont bien souvent tort d'opposer : justice contre sécurité, magistrats contre policiers ... C'est une erreur, tant ces deux sujets sont liés. Il ne peut y avoir de sécurité sans une justice efficace, et réciproquement. Côté justice, le constat est maintenant connu de tous : 93 % des Français estiment que la justice est lente, 69 % qu'elle est opaque, 68 % qu'elle est laxiste et même 53 % qu'elle est partiale

Bien sûr, il y a eu les « sucres rapides », mais ils sont venus cacher le goût amer du manque cruel de magistrats et de greffiers. Et ils ne sont venus qu'en fin de mandat Et ce n'est qu'en fin de mandat, encore, que le Président de la République aura prononcé un discours donnant sa vision de la justice, du rôle et de la responsabilité des magistrats, et ce pour inaugurer les États généraux de la justice. En outre, il est peu de dire que les deux gardes des sceaux précédents et leurs « grandes » réformes, respectivement la loi pour la confiance dans la vie politique de François Bayrou et la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice de Nicole Belloubet, n'auront pas forcément marqué les esprits. Pendant ce quinquennat, nous avons vu beaucoup de lois sur la loi, mais aucune sur l'institution judiciaire et son organisation. Certaines de ces lois permettront de rendre la justice plus plus juste : je pense au code de la justice pénale des mineurs, aux différentes lois de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, au bracelet anti-rapprochement, à l'âge en dessous duquel on ne peut consentir à un acte sexuel, à la loi sur la dignité en détention,

N'oublions pas non plus que les promesses du candidat Macron visant à renforcer les garanties d'indépendance du parquet, avec l'inscription dans la Constitution de la nomination des procureurs sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature,

tant l'enjeu est grand et les difficultés quotidiennes des magistrats importantes. Même si une bonne part de la hausse a été absorbée par le programme de construction de places de prison, cela aura permis de donner à la justice les moyens de payer ses experts et ses avocats commis d'office et d'aider à la prise en charge des victimes. de quoi la justice aurait-elle besoin ? De plus de magistrats, sans aucun doute. Sans même aller jusqu'à la moyenne européenne- nous n'avons pas forcément les mêmes pratiques -, il est clair qu'on ne peut rendre une justice sereine en siégeant dix heures d'affilée, sans pause, et en terminant à 1 heure du matin. De même, nous sommes le pays où les procureurs ont le plus de dossiers à traiter. On leur demande en sus de faire de la communication, de gérer les relations extérieures au tribunal, de discuter avec les élus et les services de l'État Jours et nuits ne suffisent plus. Et je ne parle pas des greffiers, souvent surdiplômés et sous-payés au regard des tâches qu'on leur confie. Bien évidemment, et la ministre aurait été surprise que je n'aborde pas le sujet, tout cela fonctionnerait mieux avec de bons outils informatiques- logiciels et réseaux -, mais aussi avec un peu de décentralisation. À cet égard, notre visite à Rouen, avec ma collègue Agnès Canayer, a été édifiante : des locaux vétustes et inadaptés et pas de personnel pour l'entretien Si l'on peut trouver des sucres rapides pour l'administration, trouvons-en pour la gestion des bâtiments. Faut-il que les greffiers aiment leur métier pour l'exercer dans de telles conditions ! Remercions-les

C'est une bonne mesure. Il n'est pas acceptable d'avoir des zones de non-droit dans la République et il faut entreprendre une indispensable reconquête des rues, des halls d'immeuble et des cages d'escalier.

Les victimes qui ont le courage de faire la démarche de porter plainte, et elles sont encore trop peu nombreuses, ne doivent pas rencontrer dans l'institution policière et judiciaire des difficultés supplémentaires. Attention à ne Attention à ne pas oublier, au milieu de la surenchère qu'amène souvent le thème de la sécurité, surtout en cette période, ce qui doit être au coeur de l'action de nos tribunaux, de nos commissariats et de nos gendarmeries : la victime et, à travers elle, la réparation du tort causé à la société.

Rétablir la confiance entre la police et la population : ça n'a pas marché ! Maintenir l'ordre : ça a mal marché ! Garantir les libertés publiques : ça boîte un peu ! Avec mes collègues sénatrices et sénateurs socialistes, je déplore l'état délétère des relations entre la police et nos concitoyennes et concitoyens.

Tout d'abord, la doctrine du maintien de l'ordre : il s'agissait d'une doctrine matérialisée dans un schéma discuté, parce que discutable. On en a vu les résultats : faibles. On en a vu aussi les effets : contre-productifs pour le maintien de l'ordre sur le terrain.

Ces nouvelles technologies peuvent constituer un instrument indéniable de progrès pour notre sécurité, et nos forces de l'ordre doivent en être dotées. Mais elles n'en sont pas moins intrusives. Or la protection des données personnelles et la préservation de la vie privée sont des conditions de l'État de droit,

On a dit de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi pour une sécurité globale qu'elle était un revers pour le Gouvernement. En invalidant les dispositions de l'article 47, relatif à l'usage des drones, de relatif à l'usage des caméras embarquées et de l'article 52, relatif à un délit de provocation à l'identification d'un agent, le Conseil constitutionnel souligne avant tout qu'il n'y aura pas de meilleure sécurité sans garantie de nos libertés et qu'aucune surenchère politicienne n'est justifiée.

pour chacune et chacun. La sécurité pour tous, c'est une part de la promesse républicaine. Après presque cinq ans de « marchisme », les Françaises et les Français ont pu faire un constat : en matière de sécurité, comme en d'autres matières, la République qui marche, ce n'est pas la République en marche. La législature arrive à son terme et le travail pour améliorer la sécurité de nos concitoyens est plus qu'inachevé. Madame la ministre, on ne compte plus les ministres de l'intérieur de ce quinquennat. Je sais donc que vous ne portez pas plus de responsabilité que les autres dans ce qui n'a pas fonctionné. pas fonctionné. M. Darmanin a déclaré : « Chaque Français verra plus de bleu sur le terrain en 2022 qu'en 2017 », mais une récente communication de la Cour des comptes interroge sur la faisabilité de cette promesse.

de notre responsabilité de contribuer concrètement à l'élaboration de ces budgets, car le Gouvernement agit avec les moyens que le Parlement lui confère. Nous nous sommes ainsi réjouis, l'année dernière, de la hausse historique du budget de la justice, que nous avons voté. Le budget de la justice pour 2022 s'inscrivait également dans une dynamique de hausse majeure, supérieur d'un tiers à celui de 2016. Cet effort important doit se poursuivre, car il est essentiel pour notre société. La justice de notre pays est trop souvent pointée du doigt, tenue pour responsable de l'insécurité que connaît notre société : laxiste, elle ne ferait plus respecter la loi. Nous ne souscrivons pas à ce raisonnement simpliste. Comment la justice pourrait-elle être plus ferme quand nos prisons sont pleines, et même plus que pleines, puisque le taux d'occupation moyen dans notre pays était de 114 % en octobre dernier Les maisons d'arrêt sont concernées au premier chef. Plusieurs d'entre elles dépassent les 200 %, comme celles de Nîmes ou de La Roche-sur-Yon. Cette réalité laisse imaginer les conditions de détention dans le contexte d'une pandémie toujours en cours.

Cette année, le rapporteur pour avis de commission des lois, notre collègue Alain Marc, a donné un avis favorable à l'adoption des crédits du programme pénitentiaire, alors même que des retards accumulés ne permettront une livraison de ces 7 000 places qu'en 2023.

Nous y voyons le signe d'une prise en compte des nécessités du terrain, et nous la saluons. La France compte toujours deux fois moins de juges par habitant que la moyenne européenne. La justice est pourtant au coeur du contrat social. Elle doit être efficace pour continuer d'être légitime nous ne pouvons faire l'économie d'une amélioration de ses moyens. Pour autant, les femmes et les hommes qui oeuvrent dans notre pays pour la justice et la sécurité sont pleinement mobilisés. Nous tenons à saluer leur engagement sur tous les territoires de la République. au quotidien des Français. Entre 2017 et 2022, plus de 10 500 emplois de policiers et de gendarmes auront été créés. Le président Macron a eu l'occasion de faire des annonces relatives au renforcement de la présence policière sur la voie publique. Nous croyons que cette mesure sera bénéfique à l'ensemble de nos concitoyens. Le budget que nous aurions dû examiner montrait des augmentations significatives destinées non seulement à accroître les effectifs, mais également à améliorer les locaux et les équipements de nos forces de l'ordre-

La modernisation des équipements est également essentielle. Nos forces de l'ordre, qui interviennent dans des conditions souvent très tendues, doivent pouvoir compter sur des matériels de qualité. L'ensemble de ces facteurs contribuera à améliorer les relations des forces de l'ordre et de la population. L'insécurité et le respect de la règle de droit constituent à juste titre des préoccupations majeures pour l'ensemble de nos concitoyens. L'action du Gouvernement, accompagné par le Parlement, traduit toute l'importance de la sécurité et de la justice.

madame la ministre, mes chers collègues, que de temps perdu ! Voilà ce que nous inspire l'action des ministres de la justice et de l'intérieur du quinquennat d'Emmanuel Macron en matière de sécurité et de répression de la délinquance dans notre pays.

La situation est très dégradée ; c'est la loi du plus fort qui s'impose, celle des narcotrafiquants, des islamistes radicaux, qui ont pris la place de la République dans tous les quartiers difficiles où l'on vit côte à côte, et où, demain, je crains qu'on ne vive face à face. » En quelques mots, tout est dit : le rétablissement de l'autorité de l'État est le sujet majeur auquel sont confrontées la police et la justice dans notre pays. Un retour à l'ordre qui nécessite de mettre fin à l'impunité dont bénéficient nombre de délinquants en instaurant le principe d'une sanction pénale claire, effective et immédiate. le répète, que de temps perdu au ministère de l'intérieur, qui passe du deuxième au onzième rang protocolaire avec l'épisode du ministre Castaner, empêtré dans la crise des gilets jaunes et dans des déclarations médiatiques inadaptées, voire mensongères, qui ont suscité maintes polémiques. Avec l'arrivée de Gérald Darmanin, en juillet 2020, le Parlement a pu commencer, avec trois ans de retard, à traiter les vrais problèmes, avec les lois sur la sécurité globale, le terrorisme et le renseignement. Une fois encore, que de temps perdu Madame la ministre, lors de la discussion générale sur la loi relative à la sécurité globale, le ministre déclarait vouloir organiser un continuum de sécurité. Je tiens ici à saluer l'engagement fort des maires et des élus locaux afin de toujours mieux organiser et intégrer les polices municipales à ce continuum, souvent pour pallier le défaut de présence de l'État sur le terrain en matière de sécurité. Nous avons d'ailleurs enrichi ce texte pour que la mutualisation des forces de police soit plus simple. Je veux également rappeler l'impérieuse nécessité de mieux protéger les forces de l'ordre dans un contexte d'une grande violence à l'égard de tous les fonctionnaires portant l'uniforme républicain. Quel acte manqué que la rédaction de ce fameux article 24 de la loi Sécurité globale, finalement censuré par le Conseil constitutionnel !

Je pense aussi à nos travaux sur le terrorisme et le renseignement, lois si nécessaires quand le risque terroriste demeure important, notamment avec la sortie de prison des condamnés djihadistes. Une nouvelle fois, madame la ministre, je regrette votre manque d'écoute

Finalement, nous avons manqué d'un plan-guide dans la mise en oeuvre de la politique de sécurité du pays. Je regrette que le ministre de l'intérieur n'ait pas mis en place une loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, une Loppsi, dès le début du quinquennat, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre

Pour 2022, le ministère rompt avec les pratiques antérieures en diminuant la part des dépenses de personnel au bénéfice de l'investissement et du fonctionnement. Mais les questions de gouvernance et d'heures supplémentaires sont toujours aussi mal gérées, comme le souligne, à juste titre, la Cour des comptes. Pour conclure, mes chers collègues, ce bilan de l'action du Gouvernement en matière de sécurité se déroule dans un contexte plus apaisé que celui, calamiteux, de la première partie du quinquennat. Toutefois, je le redis, seule une Loppsi serait à même de dégager et de programmer les moyens pour lutter contre la délinquance et la criminalité. Cela suppose, comme le propose notre groupe Les Républicains, de modifier la Constitution pour instaurer des peines minimales obligatoires, de mieux protéger ceux qui nous protègent et de ne plus accepter l'excuse de minorité des mineurs délinquants devant la justice. Enfin, héritiers de l'histoire de notre Haute Assemblée, nous restons soucieux de garantir les libertés fondamentales.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous faire part de mon émotion, alors que vingt-sept personnes sont mortes dans la Manche, et que cette mer, comme la Méditerranée, est en train de devenir un cimetière. La sécurité des migrants est une question d'ordre public, mais la réponse humanitaire doit primer sur les considérations sécuritaires et politiques. Si des migrants sont en danger en mer, on déploie des moyens de sauvetage ; si des migrants vivent dans des conditions indécentes, on leur donne de quoi survivre dignement. Que fait le Gouvernement dans cette histoire ? Pas grand-chose ! Enfin si, parfois, il fait, ou plutôt il laisse faire : les forces de l'ordre se permettent de harceler les réfugiés, de déchirer leurs tentes à coups de canifs et de repousser les bénévoles. Cet hiver, le drame se poursuit : plus de 97 % des expulsions de lieux de vie n'ont pas été suivies de mises à l'abri. Combien faudra-t-il de personnes mortes de froid ? Quand vingt-sept personnes meurent en une journée, que trouve à dire le ministre de l'intérieur : « c'est la faute des passeurs

en 2016, un jeune ministre de l'économie déclarait : « La sécurité n'est pas un projet politique. » Il avait raison : elle est plutôt une conséquence de nos politiques publiques, à commencer par les services publics. Bien sûr, nous saluons l'extension du budget de la justice, mais quel dommage que cette hausse soit focalisée sur la construction de nouvelles places de prison,

dégradant. Des solutions existent : plutôt que d'augmenter sans cesse le nombre de détenus, il faut développer les alternatives à la prison et créer des centres de détention semi-ouverts, sur le modèle des pays nordiques. En amont, il convient de renforcer les travailleurs sociaux, la prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiatriques ou encore le tissu associatif.

Je dois admettre qu'il m'est de plus en plus difficile d'entendre le Gouvernement se gargariser de la manière dont il traite ce qu'il appelle « la grande cause du quinquennat ». De fait, que d'occasions manquées ! Ainsi, pourquoi ne pas avoir fait modifier la définition du viol de façon à respecter nos engagements internationaux, notamment la convention d'Istanbul, pour qu'enfin le viol soit défini par l'absence de consentement de la victime ? Pourquoi ne pas avoir pris exemple sur l'Espagne en instaurant une justice et une police spécialisées qui n'aggravent pas les traumatismes

saurais conclure mon propos sans évoquer certaines promesses non tenues de ce quinquennat. Qu'en est-il de la promesse du candidat Macron de constitutionnaliser l'indépendance du parquet vis-à-vis de l'exécutif ? Qu'en est-il de sa promesse de supprimer la Cour de justice de la République ? On a plutôt eu droit à la critique d'un prétendu gouvernement des juges et au maintien au Gouvernement de ministres mis en examen. Les déclarations d'intention et la course à l'échalote sécuritaire avec la droite et l'extrême droite n'ont jamais fait une politique ; surtout, elles n'ont jamais pu protéger la justice en général ni la sécurité de qui que ce soit.

parce que cela permet d'éradiquer les trafics, de contrôler les produits et de gérer les problèmes d'addiction, qui relèvent de la santé publique. Ne serait-il pas temps de s'en inspirer, de trouver des solutions alternatives, rationnelles et pragmatiques,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à c'est le nombre de personnes qui, entre 2019 et 2020, ont été réduites de l'effectif pénitentiaire, pénitentiaire, parce que les jugements ont été moins nombreux, mais aussi parce qu'on a libéré, pour des raisons sanitaires, un grand nombre de personnes en fin de peine. Cela a-t-il créé un problème particulier dans notre société ? Non. C'est bien la preuve, madame la ministre, s'il en fallait une,

madame la ministre, mes chers collègues, c'est en ma qualité de rapporteur spécial de la commission des finances de la mission « Justice » que j'ai souhaité aujourd'hui intervenir devant vous. Afin d'être rigoureusement établi, le bilan de la justice pendant ce quinquennat mérite d'être fondé sur les indicateurs privilégiés que sont les moyens humains, financiers et matériels que lui alloue l'État. À ce titre, il serait malhonnête de ne pas reconnaître l'effort budgétaire constant accordé tout au long du quinquennat, qui a permis à l'institution judiciaire d'opérer un redressement salutaire.

Année après année, l'augmentation dynamique des crédits sur l'ensemble des cinq exercices budgétaires témoigne d'une prise en compte sérieuse par l'exécutif des défis posés par les archaïsmes de l'institution. Il est important de saluer un investissement très ambitieux pour l'ensemble de l'administration pénitentiaire. Cette dernière a bénéficié d'une importante revalorisation de ses métiers, ainsi que de la création de plus de 4 300 emplois. nombreuses et solides ont été apportées pour renforcer et faciliter l'accès du citoyen à la justice, qu'il s'agisse du portail « justice.fr », des points d'information répartis dans les territoires ou encore de la revalorisation de l'aide juridictionnelle.

En un mot, le constat laisse peu de place au doute : la justice n'a pas encore pleinement rempli les objectifs qui lui avaient été assignés pour ce quinquennat. J'en veux pour preuve la tribune désormais signée par plus de 5 000 magistrats, soit une large majorité des 9 000 juges en poste, qui fait état de la profonde indigence dans laquelle nos juges sont amenés à exercer leurs fonctions.

inlassablement ressassée par les personnels judiciaires, et fait peser sur les épaules de toute l'institution un fardeau terriblement nocif pour notre République. Pis encore, c'est un danger pour la crédibilité du système judiciaire auprès des justiciables. Comme l'a souligné le questeur Philippe Bas, nous avons systématiquement constaté, au cours des cinq dernières années, une sous-exécution des dépenses prévues en loi de finances. Ce sont au total plus de 510 millions d'euros dont la dépense, pourtant affectée en crédits de paiement, n'aura pas été concrétisée. Dans un récent rapport dressant des pistes d'amélioration pour la justice, la Cour des comptes épingle, entre autres choses, les retards accusés dans le vaste plan de transformation numérique promis par la Chancellerie, mais dont l'aboutissement vient à tarder. Ce « coeur du réacteur », selon les mots de M. le garde des sceaux, n'a pas encore été pleinement déployé, ce qui constitue aujourd'hui encore un frein notable à l'accomplissement du programme de modernisation des tribunaux : doivent en être tenues pour responsables les asymétries entre les applicatifs du ministère de la justice et ceux des ministères de l'intérieur et des finances. Je terminerai mon propos sur le point le plus sensible de ce bilan, à savoir l'inachèvement du programme pénitentiaire promis en 2017. Dès le début du quinquennat, malgré la promesse de 15 000 nouvelles places de prison, il nous a été indiqué que l'accomplissement du projet ne nécessitait non pas un mandat présidentiel, mais bel et bien deux. Voilà une remarquable preuve de confiance face aux aléas électoraux. Ce sont donc 7 000 places qui seront sorties de terre à l'horizon 2022, laissant le dramatique problème de la surpopulation carcérale dans un identique à la situation d'avant le Les points de vue divergent largement sur le nombre de places de prison à construire afin d'optimiser la sécurité des citoyens : certains avancent 20 000, d'autres davantage encore. Quel en est le nombre idéal ? Nul ne le sait. Notre priorité collective demeure toutefois de concilier le respect des droits de l'homme en détention avec la pleine exécution des peines prononcées. Je salue toutefois les deux prisons en cours de construction à Toul et à Donchery. Axés sur le travail, ces deux projets me semblent très prometteurs.

le tout couronné par des États généraux de la justice. Ces derniers, qui se veulent un grand rendez-vous oecuménique des acteurs judiciaires, ont été engagés beaucoup trop tardivement dans le quinquennat. Les efforts que nous voulons porter pour notre justice devront toujours et impérativement s'accompagner d'une réflexion de fond sur les métiers qui la structurent, ainsi que sur la juste application des sanctions prononcées. Il y va du sens de la peine et de l'indispensable confiance du justiciable dans la seule autorité détentrice de la violence légitime.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à quelques mois du terme de ce quinquennat, nous pouvons légitimement nous poser la question : quel bilan pour la justice et la sécurité ? ? La justice va mal ! Une étude menée par le Sénat dans le cadre de l'Agora de la justice démontre que 53 % des Français n'ont pas confiance dans l'institution judiciaire, même s'ils font majoritairement confiance à chacune de ses professions. Les Français reprochent à la justice sa lenteur, ainsi que son manque de transparence et d'effectivité dans l'exécution de ses décisions. En conséquence, 59 % des sondés disent ne la saisir qu'en dernier recours.

Pourquoi ces réformes et ces moyens supplémentaires ne produisent-ils pas les effets recherchés ? C'est avant tout un problème de méthode : les réformes se succèdent à grande vitesse, ce qui laisse peu de temps aux professionnels de la justice pour les assimiler. L'inflation législative et réglementaire est un facteur de paralysie de l'institution judiciaire. Certaines réformes ne font même pas l'objet d'une évaluation- ainsi de l'instauration du divorce par consentement mutuel sans recours au juge. Les difficultés sont d'autant plus réelles que ces réformes entrent souvent en vigueur avant même que les outils numériques correspondants soient à disposition des juridictions.

L'augmentation des effectifs dans les juridictions est en revanche notable. Le taux de vacance d'emploi des magistrats est désormais inférieur à 1 %. Cependant, celui des greffiers s'élève toujours à 7 %.

Si l'apport de contractuels a permis de soulager certaines juridictions, le statut et les missions de ces agents ne leur permettent pas de remplacer les magistrats et les greffiers. Une réévaluation des besoins des juridictions en magistrats professionnels doit être menée afin de faire correspondre les moyens avec les charges réelles. Une réflexion globale s'impose sur l'exercice de la profession de magistrat, et notamment sur l'équipe autour du magistrat, en particulier pour prendre en compte les nombreuses évolutions professionnelles. Enfin, la grande oubliée de ces réformes reste la justice civile, qui représente pourtant la grande majorité du contentieux, avec plus de 2 millions de décisions rendues chaque année. Il conviendrait de renforcer la déjudiciarisation, ainsi que la délégation de certaines missions à l'équipe du juge. Ces réformes, proposées par le Sénat, Sénat, permettraient de redonner confiance dans la justice du quotidien. L'effectivité de la réponse pénale constitue aussi un enjeu. Il faudrait apporter une réponse proportionnée à chaque infraction afin de prévenir la récidive et de se donner les moyens d'une véritable exécution des peines prononcées. Voilà un exemple de levier

Je veux tout d'abord rappeler que, depuis 2018, au plus près des Français, la police de sécurité du quotidien se déploie sur tous les territoires. Elle accompagne le retour de l'État là où la République a pu, par le passé, donner le sentiment de reculer sous le poids des trafics et des violences. Pour assurer ce retour, près de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires ont été recrutés pendant ce quinquennat, dont près de 1 200 dans les 62 quartiers de reconquête républicaine mis en place depuis 2018 par le ministère de l'intérieur. Toutes les circonscriptions de sécurité publique connaîtront une progression de leur effectif sur la durée du quinquennat. Leur première mission est d'intensifier la lutte contre la drogue et ses trafics.

7 837 trafics ont été démantelés, ce qui correspond à une hausse de 34 % ; 52 millions d'euros d'avoirs criminels ont été saisis. Pour être efficaces dans la lutte contre la délinquance, les trafics, la violence, nous devons prendre le mal à la racine et agir sur les facteurs de risque. Tel est l'objectif de la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024 que je porte. Cette stratégie met l'accent sur la prévention de la délinquance des mineurs dès avant l'âge de 12 ans ; sur les démarches d'aller vers les personnes les plus vulnérables pour mieux les protéger ; sur la participation de la société civile à la politique de prévention et sur le rapprochement entre la police ; sur la rénovation de la gouvernance territoriale de cette politique, en lien avec les élus locaux et l'autorité judiciaire. Cette politique de prévention ambitieuse nécessite des moyens : nous y avons consacré 70 millions d'euros cette année et nous y consacrerons 10 millions de plus l'an prochain, notamment pour accroître notre effort en faveur de la vidéoprotection des voies publiques. Pour qu'ils soient plus efficaces dans leur lutte contre la délinquance et la criminalité, nos policiers et gendarmes doivent en outre travailler dans des conditions optimales. C'est pourquoi, à la fin de l'année 2021, plus de 700 casernes et commissariats auront été modernisés et 30 000 véhicules achetés

concrets sur le terrain. L'engagement du Président de la République et du Premier ministre, à l'issue des travaux menés dans le cadre du Beauvau de la sécurité, s'est traduit par une hausse des crédits de la mission « Sécurités » de plus de 1 milliard en compte le plan de relance. Cela porte l'augmentation du budget de cette mission depuis le début du quinquennat à 2,3 milliards d'euros. Je dirai enfin un mot de la priorité absolue qu'est la lutte contre la radicalisation et le terrorisme. Nous avons commencé, dès 2017,

cadres dirigeants de l'État, en présence de M. le Premier ministre. Avec les cellules de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire (CLIR), dont les moyens juridiques ont été renforcés par la loi confortant le respect des principes de la République, nous agissons concrètement dans les territoires pour prévenir les dérives

une augmentation de 33 % depuis 2017. Face aux incivilités du quotidien, tels les rodéos motorisés, l'usage de produits stupéfiants ou les vols dans les commerces de proximité, il fallait apporter des réponses plus rapides et plus efficaces. Le développement de la justice de proximité, dont la raison d'être est précisément de répondre à ce type de délinquance, contribue à restaurer la crédibilité de la justice auprès de nos concitoyens. En apportant des réponses pénales, qui ont du sens pour les victimes et les auteurs, elle renforce notre État de droit. Nous nous sommes également concrètement attachés à renforcer les politiques pénales prioritaires : la lutte contre les violences exercées à l'encontre des forces de l'ordre, en pénalisant plus fortement leur auteur ; la lutte contre le poison que constitue le trafic de stupéfiants,

contre la haine en ligne a ainsi été créé par le garde des sceaux afin de sanctionner les discours de haine qui prospèrent sur internet. Parmi les priorités du Gouvernement en matière de justice figure bien sûr la question de la justice des mineurs. Le code de la

plus rapide pour toutes et tous. Cette réforme met aussi fin à l'empilement des mesures éducatives par la création d'une mesure éducative judiciaire unique, dont le contenu est modulable et adaptable à l'évolution du mineur.

particulièrement le budget de la protection judiciaire de la jeunesse, constitue une priorité. En deux ans, près de 95 millions d'euros supplémentaires ont permis de renforcer l'action de la protection judiciaire de la jeunesse, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur associatif habilité. La justice des mineurs, c'est aussi la protection des plus fragiles,

La mise en chantier des 7 000 premières places est d'ores et déjà lancée. En 2022, ces places seront livrées ou à un stade avancé de construction. Au total, quatorze opérations sont en cours dans toute la France,

Permettez-moi d'ailleurs de saluer ici l'esprit républicain des maires qui accueillent et soutiennent ces projets. Je pense notamment aux élus de Caen ou d'Angers. La lutte contre la radicalisation a également été marquée par un renforcement de l'arsenal législatif visant à la détection, au suivi et à l'entrave des individus susceptibles d'être radicalisés et de constituer une menace pour l'ordre public. Je tiens également à évoquer la loi du 30 juillet 2021, qui a créé la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, ou encore celle du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui a créé deux nouveaux délits aux fins de lutter contre la radicalisation violente. La prise en charge des radicalisés en établissement pénitentiaire a aussi été renforcée par la création de nouveaux quartiers d'évaluation et de prise en charge de la radicalisation. Pour répondre au sénateur Sueur et à la sénatrice

embrassent tous les thèmes d'actualité qui sont au coeur de la justice. Trois d'entre eux portent d'ores et déjà sur les moyens, les organisations et les missions des magistrats et des greffiers. C'est un exercice démocratique

tout ». Ils ajoutent : « Nous comprenons que les personnes n'aient plus confiance aujourd'hui en la justice que nous rendons, car nous sommes finalement confrontés à un dilemme intenable : juger vite mais mal, ou juger bien mais dans des délais inacceptables.

Comment redonner du sens à ces professions essentielles pour notre État de droit et pour le bien vivre ensemble, piliers de notre société ? Comment redonner leur grandeur aux politiques régaliennes dont dépendent magistrats et forces de l'ordre ? Que faire pour que ces professionnels puissent se relever face à tant de souffrance et de mépris ?

Annoncé dès 2016, cet ambitieux programme semble rencontrer des difficultés que certains jugent insurmontables. Alors que la procédure pénale numérique devait être étendue à l'ensemble des juridictions françaises en 2022, la police attend encore un outil informatique moderne devenu indispensable, car le système actuel, même dans sa dernière version la plus évoluée, est en bout de course. Un récent article du détaille les nombreuses difficultés techniques qui s'enchaînent depuis le début de ce projet et évoque un « enlisement » d'autant d'autant plus inquiétant que certains hauts responsables de la police nationale avancent que, au total, 11,7 millions d'euros seraient partis en fumée, salaires des policiers détachés compris. Madame la ministre, où en est précisément ce projet aujourd'hui

ministre déléguée. Monsieur le sénateur, le logiciel de rédaction des procédures est le coeur du système d'information de la police nationale. Vous avez raison, il est utilisé

Il devait être un outil moderne, simple à utiliser, permettant un pilotage performant. Malheureusement, le programme n'a pas répondu à ces ambitions, pour des questions de gouvernance, de priorisation et de pilotage. Face à ces difficultés majeures,

à l'échelon local quelques difficultés. Si l'État encourage, souvent très fortement, les communes à se doter de caméras de vidéoprotection, dont elles ont la responsabilité et l'initiative, l'accompagnement financier qui est censé aller de pair, est, lui, plus incertain.

Pourtant, malgré la circulaire du 5 mars 2020, qui définit les orientations triennales 2020-2022 du Gouvernement en la matière, et celle du 30 avril 2021 relative aux orientations budgétaires du fonds pour l'année 2021,

Les moyens dévolus sont trois fois inférieurs aux besoins exprimés. Que compte faire le Gouvernement sur ce sujet, qui figure parmi les préoccupations majeures des Français ? La parole

à 79,4 millions d'euros l'an prochain. De plus, 5 millions d'euros supplémentaires ont été prévus dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2021 pour financer les actions

104 victimes de trop. La dernière d'entre elles a été tuée vendredi dernier, au lendemain de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, en bas de chez elle, alors même qu'elle bénéficiait d'un téléphone grave danger.

pour que toutes les femmes en danger puissent enfin être pleinement protégées ? Quel bilan tirez-vous de la lutte contre les violences faites aux femmes ? Considérez-vous avoir fait tout ce qui était possible

qu'il nous faut combattre sans relâche tant ses conséquences sur la santé physique et psychologique sont graves. Les personnes addicts sombrent dans une immense souffrance et dans une situation de fracture humaine, marquée par la rupture sociale et familiale, la dépendance, l'isolement, voire malheureusement pis encore. Au-delà de cette souffrance, le trafic de stupéfiants constitue une menace grave pour l'ordre public et pour la cohésion de notre société. Dans certaines zones de Marseille ou de la banlieue parisienne, la République est défiée.

80 % de l'héroïne consommée dans le monde profitent aux talibans, qui dominent ce marché. Le trafic de stupéfiants est l'une des principales sources de financement des mouvements terroristes et des mafias là une autre raison de s'y attaquer. Depuis le 1 septembre dernier, les consommateurs encourent une amende forfaitaire, dont le but est d'apporter une réponse rapide à ces infractions.

À ces projets, à ces équipes prêtes à agir, s'ajoute l'action de ligues factieuses comme Génération identitaire, organisation qui se reconstruit partout en France malgré sa dissolution, sous le nom des Natifs, à Paris, ou des Remparts, à Lyon. Un sentiment d'impunité semble les habiter, puisque des militants d'extrême droite continuent de mener des actions violentes sans être inquiétés. Ainsi, dans la ville de Lyon, que je connais bien, plusieurs actions coup de poing sont restées sans réponse depuis la dissolution de Génération identitaire. L'impunité et la violence s'observent également en ligne, sur les réseaux sociaux comme sur les messageries sécurisées, où se multiplient les campagnes de harcèlement et les appels au meurtre de journalistes, de politiques, d'immigrés, de juifs et de musulmans. La violence est aussi dans certains médias, où toutes les digues ont sauté. On peut aujourd'hui lire les tribunes de généraux factieux ou de responsables politiques complotistes, appelant tout simplement à l'insurrection armée. On peut aussi entendre les inspirateurs de terroristes d'extrême droite exposer leurs théories criminelles en direct sur les plateaux de télévision. Ce qui se passe dans notre pays est plus qu'inquiétant. Pourtant, du côté du Gouvernement, la réponse reste timide. On salue le travail des services de renseignement, on se félicite des attentats déjoués, mais on manque d'une approche globale.

Madame la ministre, ma question est simple : votre gouvernement va-t-il enfin prendre la mesure de la menace que l'extrême droite fait peser sur notre sécurité et mettre fin à l'impunité dont jouissent ces militants ? La parole est à Mme la ministre

de tous ces discours en ligne, y compris, bien entendu, quand ils viennent de l'extrême droite. Toutes ces mesures, et bien d'autres encore, démontrent l'engagement du Gouvernement pour lutter contre les menaces violentes émanant de l'extrême droite. Nous en